accompagné d’une délégation sénatoriale composée des présidents des groupes politiques et des présidents des groupes d’amitié France Israël et France Palestine. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du Bureau du Sénat, j’appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Mme Marie Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ma question s’adresse et Républicain. Ma question s’adresse à Mme la Première ministre. Madame la Première Ministre, vous vous seriez vantée, il y a peu, d’avoir réussi en quelques jours ce que Gérald Darmanin n’avait pas su faire en un an. Mais à quel prix ! Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front national. Au soir de son élection face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d’être un barrage contre le Front national et ses idées. Il ajoutait : « J’ai conscience que ce vote m’oblige. » Aujourd’hui, l’extrême droite n’a plus besoin d’être élue : vous appliquez son programme et faites vôtre la préférence nationale. Vous affirmez pourtant que ce projet de loi est conforme à vos valeurs. Madame la première ministre, supprimer l’aide médicale de l’État (AME), est ce conforme à vos valeurs ? Priver des étrangers en situation régulière de prestations sociales, est ce conforme à vos valeurs ? Fermer la porte de nos universités aux étudiants étrangers, est ce conforme à vos valeurs ? Écarter les étrangers des dispositifs d’hébergement d’urgence, est ce conforme à vos valeurs ? Soutenir un texte dont plus de vingt mesures sont inconstitutionnelles, est ce conforme à vos valeurs ?

a mêlé ses voix à celles du Rassemblement national pour ne pas discuter du texte. Vous n’obtenez que le fruit de votre petite politique politicienne. Mais nous, hier, nous avons su faire adopter un texte,

réplique. le ministre, je connais bien ce texte : j’ai passé quatorze heures en commission mixte paritaire. Si vous ne croyez pas ce que je viens de vous dire ou si vous pensez que c’est un mensonge, écoutez les présidents d’universités et les responsables de grandes écoles

Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre ! » Il faut conclure ! C’est sans doute aujourd’hui ce que vous êtes en train de faire.

fracturé notre République en instrumentalisant les colères populaires nées des multiples crises que nous traversons et en désignant les étrangers comme boucs émissaires. Alors que des millions de nos concitoyens ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, pensant faire barrage aux idées de l’extrême droite, ils découvrent ce matin le tapis rouge que vous lui avez déroulé avec cette loi de stigmatisation et de paupérisation de tous les étrangers : durcissement du regroupement familial, du droit du sol, des conditions d’accueil des étudiants instauration de quotas ; rétablissement du délit de séjour irrégulier… Cette commission mixte paritaire, directement pilotée par l’Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs, est en fait un nouvel accord de gouvernement entre vous et la majorité de droite radicalisée sur un programme lepéniste des années 1980. Ne vous offusquez pas, chers collègues, car l’instauration de la préférence nationale pour les prestations sociales, c’est bien du Jean Marie Le Pen ! J’alerte nos compatriotes qui pensent que leur situation personnelle peut s’améliorer avec la préférence nationale : qu’ils se souviennent bien que le recul des droits des étrangers précède toujours le recul des droits de toutes et de tous. Et vous savez de quoi vous parlez ! Cette loi est une souillure pour notre pays. La France ne sera jamais une nation ethnique elle reste une nation politique, qui repose sur des valeurs – liberté, égalité, fraternité – et sur une longue tradition d’accueil. Elle s’est construite aussi avec les vagues d’immigration, ne vous en déplaise Madame la Première ministre, renoncez à promulguer cette loi et n’inscrivez pas à l’ordre du jour la suppression de l’aide médicale de l’État l’année même où notre pays va faire entrer au Panthéon

Ma question s’adresse à Mme la Première ministre. Récemment, la presse a fait état de l’enrichissement spectaculaire de l’ancien ministre du numérique Cédric O, entré au capital de la société Mistral AI,

Comment est il possible qu’un ancien ministre, parti pantoufler dans une entreprise qui défend forcément ses intérêts propres et ceux de ses actionnaires, puisse siéger dans ce comité, censé éclairer l’action publique dans ce domaine stratégique pour la France ?

sous l’impulsion du Président de la République, c’est la France qui porte avec le plus d’ardeur le principe de souveraineté numérique en Europe, auquel vous êtes si attachée. C’est la France qui a convaincu ses partenaires européens que nous ne sommes pas condamnés à être des vassaux des Gafam. C’est encore la France qui a soutenu pour le, les réseaux sociaux et les places de marché l’adoption des règles les plus exigeantes de l’histoire récente pour mettre fin à la suprématie des géants du numérique. Avec Bruno le Maire,… Où est il ? … nous avons adopté, sur l’intelligence artificielle, une position radicalement favorable à l’innovation européenne. Parce que nous avons pris un train de retard sur les Gafam, il nous faut désormais avoir un train d’avance sur l’intelligence artificielle afin de nous affranchir de leur emprise. Parce que nous savons que la domination technologique précède la domination économique et politique, nous ne pouvons passer à côté de cette révolution numérique. La meilleure protection que nous puissions offrir à nos concitoyens, à nos auteurs, à nos artistes et à nos journalistes est de concevoir en Europe des intelligences artificielles forgées au feu de nos grands principes. Aussi, sous l’autorité de la Première ministre, nous poursuivrons les discussions dans cet esprit en veillant attentivement à préserver les capacités d’innovation européennes. Nous n’avons que faire des intérêts particuliers : seul nous importe l’intérêt national

du juste équilibre entre soutien à l’innovation et respect de nos fondamentaux ? Le secteur de la création et des médias notamment, très inquiet comme nous tous sur ces travées, compte sur vous. La parole

Madame la Première ministre, nous nous réveillons tous un peu groggy, inquiets et en colère. Le texte sur l’immigration va laisser des traces,

la recherche à tout prix, quoi qu’il en coûte, d’un texte au cœur de jeux politiciens a donc mené à l’adoption par les deux chambres d’un texte de droite fondé sur les programmes et les slogans de l’extrême droite. Plus que la fin du « en même temps », le texte marque l’affirmation réelle de l’alliance majoritaire du Gouvernement avec Les Républicains, l’affirmation du « tout à droite Quels sont les prétendus constats et analyses qui structurent ce texte ? Nous avons assisté à la construction d’une politique publique sur des faits alternatifs, sur une réalité virtuelle. La majorité et le Gouvernement ont hier validé des théories fantasmées : celles des appels d’air, des submersions migratoires, d’un système social dont profiteraient les étrangers au point de ruiner la France, celles de l’essentialisation de l’étranger comme un danger, du lien entre immigré et terroriste. Tous ces mythes ont pourtant été battus en brèche par les faits, comme le démontrent notamment les travaux du Collège de France. Madame la Première ministre, assumez vous d’avoir fondé le débat public sur des affabulations et sur des mensonges ?

l’acte majeur de notre vie démocratique, le Parlement a été piétiné tout au long de la procédure. À l’Assemblée nationale, aucun amendement de la partie relative aux recettes n’a été discuté en séance publique – aucun ni en première ni en nouvelle lecture. Vous utilisez le 49.3 non pas pour mettre un terme aux débats, mais pour empêcher tout débat. Au Sénat, nous avons passé plus de 150 heures sérieuses, constructives, responsables, à examiner ce texte. Nous avons fait des propositions, nous avons voté des économies.

En snobant le Parlement, vous vous moquez des Français. Pourquoi tant de mépris ? Que – qui – craignez vous ? Combien de temps encore allez vous ignorer le Parlement pour l’examen du budget de la France ?

Depuis près d’une décennie maintenant, nos élus se retrouvent confrontés à des blocages grandissants dès lors qu’ils cherchent à souscrire une assurance pour leur collectivité. C’est vrai ! En effet, de nombreux maires, adjoints, conseillers municipaux, directeurs généraux des services (DGS) me font quotidiennement part de leurs difficultés à cet égard et, souvent, de leur amertume vis à vis de leur assureur historique. Je crois d’ailleurs pouvoir associer de manière transpartisane bon nombre de mes collègues sénateurs à ce constat, tant cette sollicitation est devenue récurrente et malheureusement banale.

La situation est connue et plusieurs constats s’imposent à nous. Ne rejetons la faute ni sur les assureurs ni sur l’État. Nous savons que, sur le long terme, les assureurs ne pourront pas agir seuls et que l’État ne pourra pas intervenir sans les assureurs. Ce sujet est latent et ne fait que s’aggraver d’année en année.

Croire en l’apaisement social à court et moyen termes et à une diminution des catastrophes naturelles est, sinon une chimère, à tout le moins une hypothèse extrêmement risquée. Considérer que les communes pourront s’auto assurer pour tous les sinistres sans causer de déroutes financières et démocratiques majeures, alors que leur budget est déjà extrêmement contraint, est tout aussi illusoire.,

En politique comme en assurances, la véritable grandeur réside dans la capacité à protéger et à assumer la responsabilité. C’est en effet en anticipant les risques que nous assurons un avenir sûr pour notre société. Nos maires n’attendent qu’une chose : être réassurés, pour être rassurés

Nous voilà rassurés ! Un certain nombre d’événements récents, notamment l’épisode de violences urbaines au début du mois de juillet dernier, ont de nouveau démontré l’absolue fragilité du système d’assurances de nos collectivités territoriales.

énergétique. Madame la ministre, je veux vous interroger sur la mise en concurrence des concessions des barrages hydroélectriques imposée par la Commission européenne à la France depuis une mise en demeure du 22 octobre L’hydroélectricité, énergie renouvelable, flexible et stockable, que nous connaissons bien en Corrèze, demande de la visibilité et de la stabilité. de transport d’électricité (RTE), rappelle que son développement constitue une ressource indispensable, quel que soit notre futur mix énergétique. Ce sont ainsi près de 5 gigawatts supplémentaires qui doivent être développés à l’horizon de 2050.

a annoncé vouloir promouvoir l’hydroélectricité en proposant « un nouveau cadre législatif qui permettra de relancer rapidement les investissements dans nos barrages

enfin libérer les investissements pour nos barrages, sans passer par une mise en concurrence ? Est ce possible en passant d’un régime de concession à un régime d’autorisation d’exploitation ?

vous avez raison, les barrages hydroélectriques font partie de notre patrimoine national. Ils sont d’abord la fierté de nos vallées et matérialisent la France des bâtisseurs. Je le dis sans ambages : je suis engagée sans aucune réserve dans le développement de l’énergie hydroélectrique. Aujourd’hui, la France compte 2 600 installations hydroélectriques : cela représente 26 gigawatts. C’est notre première énergie renouvelable : celle ci est pilotable et permet de renforcer la résilience de notre système électrique. Elle sera donc essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques et pour sécuriser notre approvisionnement en énergie. Comme vous le rappelez, monsieur le sénateur, la Commission européenne a engagé un précontentieux contre la France, ce qui bloque un certain nombre d’investissements dans des concessions aujourd’hui échues. C’est pourquoi je travaille sur plusieurs pistes, qui doivent répondre à cinq objectifs clairs. Premièrement, relancer rapidement les projets de développement actuellement bloqués, notamment des projets de Step. Deuxièmement, garder la pleine maîtrise de notre parc hydroélectrique en évitant les mises en concurrence.

faire en sorte que l’ensemble des bénéfices résultant de l’exploitation des concessions bénéficient à la collectivité. Cinquièmement, disposer de contrats souples avec des possibilités de modifications

d’exploitation, laquelle permet une transmission du patrimoine aux opérateurs avec un cahier des charges très sécurisé pour permettre à la collectivité locale de reprendre la main. Il faut conclure, madame la ministre. Certains

Madame la ministre, depuis cette mise en demeure européenne, nous avons perdu dix ans dans le financement de modernisations permettant l’augmentation de production des barrages et la mise en place de Step. Et voilà ! Sans prorogation des concessions, EDF ne pouvait en effet pas investir.

et que cette absence de réponse créait chez les individus concernés un sentiment d’impunité inacceptable. C’est vrai. Que demandent ces maires ? Ils demandent justice pour ne plus être seuls, en première ligne, face à des individus qui se considèrent au dessus des lois.

Notre démocratie est vivante, la démocratie locale particulièrement. La violence n’y aura jamais sa place : il n’y a de place, et cette place est grande, que pour la loi, le débat démocratique et le suffrage universel.

Le climat doit s’apaiser ; à défaut, les hussards bleu blanc rouge de la République tomberont les uns après les autres, ce qui affaiblirait notre démocratie locale. Être élu de la République, c’est un engagement, pas un sacrifice. Monsieur le garde des sceaux, que répondez vous à ces maires qui demandent, dans les Alpes de Haute Provence comme ailleurs, des réponses pénales plus adaptées

s’en prendre à un élu, c’est s’en prendre à la République. C’est pourquoi j’ai placé la justice de proximité au cœur de mon action. Vous avez d’ailleurs rappelé

notamment, de 1 700 point justice. Enfin, et bien sûr, elle suppose une réponse pénale implacable contre tous ceux qui s’en prennent à nos élus. Cette politique claire doit être déclinée partout – je dis bien : partout ! – sur le territoire. J’ai reçu l’appel des maires que vous relayez, monsieur le sénateur, et je vous remercie de le faire. Les élus doivent évidemment être entendus et

prochain dans votre département, afin que le dialogue reprenne, car la sécurité de nos compatriotes impose que tous les acteurs se mettent autour de la table et que chacun fasse de son mieux pour que vive notre pacte républicain. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour le groupe Les Républicains.

la sénatrice, vous interrogez Mme la Première ministre sur le dialogue social, notamment sur les suites que nous entendons donner aux discussions des partenaires sociaux relatives à la convention de gestion de l’Unédic.

Ces engagements ont été tenus et en cela la lettre de cadrage a été respectée. Nous avons aussi demandé aux partenaires sociaux de respecter une trajectoire financière. La convention qu’ils nous présentent respecte cette trajectoire en prévoyant notamment une économie sur ce que l’on appelle parfois la filière seniors de l’Unédic. Nous avons enfin demandé aux partenaires sociaux de tenir compte de la de tenir compte de la réforme des retraites et de modifier les deux bornes d’âge à partir desquelles la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi considérés comme des seniors, c’est à dire 53 ans et 55 ans, sera décalée de deux ans, conformément à la réforme des retraites. De même, nous souhaitions que la filière de maintien des droits, qui commencent à 62 ans, soit décalée à 64 ans. Les économies inscrites par les partenaires sociaux dans le projet de convention correspondent à ces éléments. En revanche, les partenaires sociaux nous ont dit envisager l’inscription de ces propositions et de cette modification des bornes d’âge dans l’accord national interprofessionnel sur les seniors dont nous leur avons confié la discussion jusqu’au 15 mars prochain.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, ma question s’adresse à Mme la ministre de la transition énergétique. La COP28 s’est achevée la semaine dernière sur une tonalité en demi teinte en l’absence du vote des États insulaires, pourtant concernés au plus haut point

aurait constitué un premier pas significatif vers une réelle sortie des énergies fossiles, au moment où de nouveaux forages sont à l’ordre du jour en mer du Nord, au Canada et même en Gironde Pour que les actifs fossiles deviennent des actifs échoués, il faut que les pays développés montrent la voie en s’interrogeant sur les subventions publiques accordées aux combustibles fossiles, qui ont atteint un niveau record. Quel est le calendrier de suppression des niches fiscales favorables aux énergies fossiles ? Alors que l’Agence internationale de l’énergie nous rappelle que la trajectoire de 1,5 degré est encore atteignable, défendrez vous dans notre future contribution nationale une régulation de nature financière d’enrayer la prolifération des énergies fossiles ? Doit on voir dans la participation de la France à des groupes de travail sur la finance climatique une volonté du Gouvernement de mettre en place une législation bancaire contraignante et audacieuse ?

objectifs : pic des émissions en 2025, baisse de 43 % des émissions en 2030 et neutralité carbone en 2050. Tout cela figure dans ce texte.

Est il bien raisonnable, monsieur le garde des sceaux, qu’avant même le début des travaux de ladite commission et alors qu’aucune version du texte ne pouvait alors être tenue pour certaine, des magistrats se mettent en grève au motif que certaines dispositions qui ne leur conviendraient pas puissent figurer dans un projet de loi ?

pour le législateur d’exercer sa difficile tâche en toute indépendance, hors de toute pression politique ou autre. Très bien

critiquaient le texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui revenait en partie sur la simplification du contentieux des étrangers. Le texte voté hier est revenu à la rédaction du Sénat, qui est conforme aux recommandations du Conseil d’État et permet une réelle simplification

il sera soumis au Conseil constitutionnel ; une fois promulgué, il deviendra la loi de la République. Et les magistrats, qu’ils soient administratifs ou judiciaires,

Madame la ministre, ce lundi, le procès de Jimmy Lai s’est ouvert à Hong Kong. Jimmy Lai, ce Hongkongais francophile qui a choisi la France pour s’y marier, est le fondateur du quotidien hongkongais hongkongais indépendant, fermé en 2021 pour avoir soutenu les manifestations prodémocratie. Âgé de 76 ans, le lauréat du prix pour la liberté de la presse décerné par Reporters sans Frontières a déjà passé trois années dans une prison de haute sécurité, sur le fondement d’accusations montées de toutes pièces. Aujourd’hui accusé de sédition et de « conspiration avec des forces étrangères », il risque la perpétuité en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 pour faire taire la contestation à Hong Kong. Pékin a décidé de transgresser ses engagements internationaux, pris lors de la rétrocession de Hong Kong. Xi Jinping, c’est la liberté d’oppression Jimmy Lai, c’est la liberté d’expression. Citoyen britannique, Jimmy Lai aurait pu quitter Hong Kong. Malgré les périls imminents, il n’a jamais fléchi dans son engagement en faveur des droits fondamentaux et de la démocratie. Alors que s’ouvrait son procès, plusieurs pays ont appelé publiquement les autorités de Hong Kong à mettre fin aux poursuites intentées contre Jimmy Lai et à le libérer. Madame la ministre, quelle est la position de la France ?

d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, retenue par une réunion sur la situation au Proche Orient avec nos partenaires. La situation des droits de l’homme à Hong Kong est très préoccupante. Trois ans après l’adoption de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, le bilan est sans appel : nous assistons à une inquiétante érosion de la démocratie et à un démantèlement systématique des droits et des libertés.

de s’y rendre, conformément à l’approche de l’Union européenne consistant à soutenir les militants prodémocratie et les défenseurs des droits à Hong Kong.

Nous continuerons de marquer l’importance du respect de l’État de droit à Hong Kong dans nos échanges bilatéraux avec la Chine. La

le parti communiste chinois est devenu le deuxième régime, après celui des nazis, à avoir laissé mourir un prix Nobel de la paix dans ses prisons. Le régime de Xi Jinping est sans états d’âme. Mes chers collègues, unissons nos appels pour libérer Jimmy Lai et le sauver !

pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, le Président de la République a annoncé récemment la création d’un conseil scientifique, ou plutôt d’un conseil présidentiel de la science – ce n’est pas tout à fait la même chose –, composé de douze éminents spécialistes dans leur domaine de référence. de référence. On peut comprendre l’intérêt de s’appuyer sur les avis éclairés de scientifiques pour prendre des décisions stratégiques qui engagent l’avenir du pays pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais on peut aussi s’interroger sur le rôle et le fonctionnement effectif de ce prochain conseil, et même sur l’attention que voudra bien lui accorder un Président de la République dont la capacité d’écoute n’est pas la première des qualités. des qualités. Monsieur le ministre, ne craignez vous pas que ce nouveau conseil ne se transforme en l’un de ces comités Théodule dont notre pays a le secret et dont l’efficacité est souvent inversement proportionnelle à la médiatisation ?

À l’heure où nous envisageons d’explorer Mars, il serait peut être temps de faire atterrir Jupiter

et Républicain. Monsieur le ministre du travail, je reviens une nouvelle fois vers vous au sujet des travailleurs de plateformes. Le temps passe et le champ de

Elle m’avait répondu que le temps législatif européen était long. Deux ans après, nous y sommes. Un vote aura lieu vendredi matin sur le compromis entre Parlement européen et Conseil. Monsieur le ministre, la France soutiendra t elle cette harmonisation sociale par le haut ?

prises au ministère du travail pour organiser les élections permettant la représentation des travailleurs de plateformes. Le modèle que nous avons mis en place fonctionne. Pas plus tard qu’hier, trois accords ont été proposés, permettant, par exemple, de relever le prix minimal de course, de garantir un revenu horaire et kilométrique, et d’assurer une plus grande liberté tant pour les chauffeurs que pour les livreurs dans le choix des courses qu’ils veulent ou ne veulent pas effectuer. Depuis le début de l’année, une dizaine d’accords ont été soumis à discussion, au vote et à signature. La directive qui sera proposée au Comité des représentants permanents vendredi concernant les travailleurs de plateformes est issue des trilogues entre le Parlement, la Présidence espagnole et le Conseil des ministres européens du travail. Elle est très différente du projet du Conseil. Le du projet du Conseil. Le 12 juin dernier, la France a soutenu l’initiative du Conseil européen des ministres au travail et nous avons voté en faveur de la directive. Nous avions dit

Vous feriez mieux de la dissoudre. D’ailleurs, nous n’en aurons plus besoin si vous votez pour la directive, ce qui ne semble être le cas. Avec Emmanuel Macron, vous vous glorifiez d’être les seuls détenteurs détenteurs du flambeau européen, mais, vendredi, c’est bien vous qui porterez un coup fatal à la construction d’un socle de droits sociaux pour des travailleurs qui en sont dépourvus. Vous refusez que l’Europe soit synonyme de progrès social ! Vous confirmez être l’État au service du marché Vous abîmez la valeur du travail et organisez la précarité des jeunes générations ! Vous abandonnez les travailleurs et les livrez en pâture au capitalisme le plus sordide, comme hier vous abandonniez les sujets migratoires à l’extrême droite Cessez votre « en même temps » du pire et revenez aux fondamentaux républicains ! La parole est à Mme Martine Berthet, pour le groupe Les Républicains.

doit devenir l’unique interlocuteur des entreprises pour déclarer leur création, les modifications de leur situation ou la cessation de leur activité. Ces dernières redoutent désormais la fin de toutes les procédures transitoires, alors que de très nombreux dysfonctionnements perdurent. Le guichet unique ne traite actuellement que 36 % des demandes de modification et 20 % des cessations d’activité ne sont toujours pas enregistrées. Par ailleurs, les procédures effectuées par cette voie censée simplifier les démarches se révèlent bien plus complexes et fastidieuses, avec des délais de traitement qui explosent, là où il fallait

pour garantir une mise en œuvre correcte du guichet unique, madame la ministre ? Dans l’attente, la prolongation de la procédure de secours est elle bien envisagée dès le 1 janvier 2024

nécessite des ajustements et des améliorations. Nous y sommes attentifs, pour que nos entreprises puissent plus facilement déposer leurs formalités de création, de modification ou de cessation d’activité. La situation, si elle n’est toujours pas satisfaisante aujourd’hui, s’est améliorée depuis le début de l’année. Vous le savez, tous les types de formalités sont désormais disponibles sur le guichet. millions de déclarations ont été déposées depuis le début de l’année. Au 30 novembre 2023, on comptait depuis l’ouverture du guichet un flux de plus de 12 000 formalités par jour, avec un objectif de 20 000 formalités par jour. Le guichet unique reçoit donc 100 % des formalités de création d’entreprises, et plus de 80 % des autres formalités. Il est monté en puissance et en qualité, comme en attestent les chiffres que je viens de partager avec vous, pour les formalités de création, de dépôt, de cessation ou de modifications. L’enjeu est désormais de garantir la continuité et l’amélioration du service pour tous les déclarants, notamment dans les modifications de société,

Mais l’incrédulité a laissé place à la stupéfaction quand j’ai appris que ni le président de la Fédération nationale des chasseurs ni le syndicat des armuriers n’en avaient été informés. Un bar tabac est il vraiment le lieu le plus approprié pour vendre des munitions pour armes à feu ? Aux côtés de boissons, jeux de hasard, journaux et d’une multitude d’autres articles, doit on vraiment trouver des cartouches qui ne soient pas de cigarettes ? Par ailleurs, la vente des munitions ne va t elle pas exposer les buralistes à de nouveaux dangers ? De nombreux tabacs ont été attaqués et pillés durant les émeutes urbaines. Que se serait il passé si les voyous avaient en plus volé les munitions ? Après seulement deux jours de formation, les buralistes seront ils vraiment à même de conseiller les chasseurs ? Il y a là un vrai risque de sécurité

Au final, madame la ministre, pour que cela ne ressemble pas au scénario d’un mauvais film, pouvez vous nous rassurer pour que la sécurité de chacun reste garantie ? La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24 janvier 2022 prévoyait également des mesures en matière de ventes d’armes, notamment pour mettre en application des dispositions de la directive européenne de 2021 relative au commerce des armes à feu. Un décret du 3 juillet 2023, pris en application de cette loi, a réformé la délivrance des certificats professionnels nécessaires pour la vente de munitions. Deux points sont à souligner : d’une part, les buralistes devront suivre une formation

Pour nous, le lien formel avec un armurier référent garantit l’approvisionnement en munitions et la qualité de service de ce commerce de détail, particulièrement attendu dans les départements ruraux,

Une fois encore, madame la ministre, vous auriez été bien avisée de dialoguer avec le Parlement : nous avons ici des idées, et surtout la capacité de les travailler pour en tirer le meilleur

La séance est suspendue.

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié. Personne ne demande la parole ?… Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte. L’ordre

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables

et structurant de nos relations bilatérales, tant pour soutenir le dynamisme économique de la région que pour faciliter le quotidien des travailleurs frontaliers. Les sénateurs représentant les départements frontaliers de nos voisins européens ne me contrediront pas sur ce point. En 2018, date du premier accord entre nos deux pays, 90 000 travailleurs frontaliers traversaient chaque jour la frontière par la route ou le rail. Nous nous étions alors accordés sur le cofinancement d’infrastructures de transports collectifs pour augmenter la capacité des lignes ferroviaires et promouvoir une mobilité plus durable entre la France et le Luxembourg. En 2023, 122 0000 Français traversent chaque jour la frontière luxembourgeoise. Ce nombre, en constante augmentation, pourrait doubler à l’horizon de 2050. Les axes routiers et ferroviaires sont régulièrement saturés. vivre… Très difficile ! … pour les travailleurs frontaliers, contribue en outre à accentuer l’impact environnemental du transport routier. Dans ce contexte, il est essentiel de poursuivre le renforcement de la coopération entre la France et le Luxembourg sur les mobilités, afin de réduire les fortes nuisances que cette situation produit pour nos concitoyens. C’est pourquoi, lors de la commission intergouvernementale de 2021, nous nous sommes engagés avec les autorités luxembourgeoises à augmenter, chacun à hauteur de 110 millions d’euros, nos contributions en faveur de notre enveloppe globale dédiée à la mobilité. L’objectif, vous l’aurez compris, est de renforcer les actions déjà engagées sur la base du protocole de 2018. Très concrètement, ces nouveaux financements permettront de poursuivre le programme d’investissements ferroviaires sur la voie entre Metz et Luxembourg, engagé dans le cadre de l’accord de 2018. Les travaux prévus par ce dernier et son avenant de 2021 permettront de passer, sur la voie entre Metz et Luxembourg, de 8 000 places assises par jour et par sens à 14 000 places en 2025 et jusqu’à 22 000 places à l’horizon 2028 2030. Les actions soutenues conjointement avec le Luxembourg permettront d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens en offrant des solutions de mobilité alternatives à l’usage encore trop répandu de la voiture individuelle par les frontaliers. Elles s’inscrivent aussi en cohérence avec nos engagements environnementaux, qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens où qu’ils se trouvent.

et le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui proposé à votre approbation. La parole

quelque 123 000 Français traversent quotidiennement la frontière luxembourgeoise pour se rendre à leur travail. Leur nombre ne cesse de croître, puisque l’on compte chaque année 3 000 travailleurs frontaliers supplémentaires. Cette situation pose inévitablement un problème de transport sur notre territoire : l’autoroute A31 est régulièrement congestionnée aux heures de pointe et l’axe ferroviaire Metz Thionville Luxembourg est confronté à des incidents fréquents, ainsi qu’à des irrégularités de service, liés à la saturation de la ligne. Pour répondre à ces difficultés, un schéma de mobilité transfrontalière a été adopté en 2009. Il vise à développer une offre de transports collectifs comme alternative à la voiture individuelle. La part du train et du bus doit ainsi progressivement passer de 10 % à 25 % d’ici à 2030. Les études conduites sur le sujet ont donné lieu notamment à la conclusion d’un protocole d’accord, dont l’approbation a été autorisée par le Parlement voilà quatre ans. Ce texte tend à mettre en œuvre aux horizons 2024 et 2030 une politique de transports multimodale et concertée entre les deux parties s’inscrivant dans la perspective du développement durable. Dans le domaine ferroviaire, les aménagements envisagés visent à tripler le nombre de voyageurs quotidiens, grâce notamment à la création de parkings relais, à l’allongement des quais dans huit gares et au doublement des places assises dans les trains express régionaux (TER) aux heures de pointe. Dans le domaine routier, l’objectif est de développer des lignes de cars transfrontaliers, ainsi que le covoiturage. Pour ce faire, les infrastructures routières existantes doivent être adaptées : côté français, l’autoroute A31 doit être élargie à trois voies entre le nord de Thionville et la frontière tandis qu’un contournement de Thionville par l’ouest doit être créé ; côté luxembourgeois, une troisième voie de circulation est prévue sur l’autoroute A3, ainsi que l’aménagement de sa bande d’arrêt d’urgence en voie réservée aux cars. Aux termes du protocole d’accord, 220 millions d’euros ont été alloués au volet ferroviaire du projet et près de 10 millions d’euros au volet routier, avec un financement à parité par la France et le Luxembourg. Quatre ans après l’approbation de ce premier texte, la plupart des aménagements ferroviaires prévus pour 2024 ont été réalisés ou le seront prochainement avec un très léger retard. La région Grand Est devra ensuite acquérir des trains à trois unités mobiles, contre deux actuellement, et construire un centre de maintenance à Montigny lès Metz pour ces nouvelles voitures, puis revoir la fréquence de passage des trains en lien avec la SNCF, afin de passer de cinq à huit TER par heure en période de pointe. En revanche, dans le domaine routier, aucune avancée ne s’est concrétisée pour le moment, au grand dam des Lorrains qui utilisent fréquemment l’autoroute A31. Seule une séquence de concertation s’est tenue il y a un an pour éclairer l’État dans le choix du tracé du contournement de Thionville. D’après l’ de la direction de la direction interdépartementale des routes Est, la situation s’est particulièrement aggravée depuis 2017. Ainsi, en l’espace de cinq ans, le temps de parcours des frontaliers s’est allongé de moitié aux heures de pointe. L’avenant au protocole d’accord soumis à notre examen vise à prolonger les objectifs fixés en 2018, c’est à dire accompagner l’augmentation des flux entre la France et le Luxembourg tout en renforçant les mobilités durables. Le Premier ministre luxembourgeois a annoncé une nouvelle contribution financière de 115 millions d’euros pour les infrastructures d’intérêt commun. Cette participation s’accompagnera d’une contribution française identique et permettra de compléter le programme d’investissements. Mes chers collègues, ce texte test essentiel pour répondre aux difficultés de mobilité quotidiennes rencontrées par nos concitoyens frontaliers. Néanmoins, au regard de l’augmentation croissante du nombre de Français travaillant au Luxembourg

En tant que conseiller régional de la région Grand Est – je salue d’ailleurs ma collègue Véronique Guillotin, ici présente –, je puis vous assurer que cette question est au cœur des préoccupations de notre région, qui finance la moitié des investissements réalisés, et même l’intégralité du futur centre de maintenance de Montigny lès Metz. Le Gouvernement a, lui aussi, pris la mesure du problème, comme en témoignent la conclusion de ces deux accords bilatéraux et la participation de l’État au financement des infrastructures.

Le transport routier est donc une solution incontournable, à condition de développer les lignes de cars et de favoriser le covoiturage. Je précise à cet égard que, depuis 2010, les émissions d’oxyde d’azote ont baissé de près de moitié dans la région, grâce aux seuls progrès technologiques réalisés sur les moteurs des véhicules, alors même que le trafic routier n’a cessé d’augmenter. Le développement du télétravail peut également constituer une réponse satisfaisante, puisqu’elle peut être mise en œuvre rapidement pour certains métiers. À ce titre, la France vient de signer l’accord européen rehaussant le seuil social de 25 % à 49 % du temps de travail. Sur le plan bilatéral, la France a accepté l’an dernier de relever le seuil de tolérance fiscale à trente quatre jours par an, contre vingt neuf jours précédemment. Au delà, le travailleur frontalier sera, bien évidemment, imposé en France. Pour augmenter plus significativement ce seuil, une solution pérenne devra toutefois être trouvée sur le partage de l’impôt sur le revenu du télétravail,

En clair, il faudra que le Grand Duché accepte de rétrocéder à la France une partie des impôts des travailleurs frontaliers, comme il le fait déjà avec la Belgique. En effet, le Luxembourg a perçu 48 millions d’euros de compensation fiscale en 2022, au titre des 50 000 travailleurs belges qui y occupent un emploi. Pour rappel, la France compte actuellement 123 000 travailleurs frontaliers, soit le quart de la population active du Grand Duché. En 2018, Xavier Bettel, alors Premier ministre du Luxembourg, déclarait qu’il ne souhaitait pas que cet argent serve à « payer la décoration de Noël » en France et qu’il préférait investir dans la qualité de vie des frontaliers. En tant qu’ancien maire de Rixheim, commune du Haut Rhin proche de la Suisse, je peux pourtant vous assurer que les communes frontalières utilisent cet argent à bon escient, afin d’entretenir les routes empruntées par les frontaliers eux mêmes ou encore d’agrandir les parkings des gares qu’ils utilisent. Le mode de fonctionnement actuel n’est pas acceptable, puisqu’il conditionne l’avancement des différents projets à la bonne volonté du Luxembourg, alors qu’il y va de ses intérêts. Dès lors, il serait utile de réfléchir à une alternative, par exemple par le montant de la rétrocession fiscale des projets décidés par la commission intergouvernementale franco luxembourgeoise. Il pourrait s’agir de projets d’infrastructures ou de financement de la formation professionnelle, dans la mesure où une partie des personnes formées en France grâce aux crédits de la région vont exercer leur profession de l’autre côté de la frontière. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce projet de loi, qui tend à résoudre ce problème persistant et à améliorer le quotidien de nombreux Français résidant près de la frontière luxembourgeoise. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la liaison Metz Thionville Luxembourg est sans doute la plus empruntée du corridor européen mer du Nord Méditerranée, et on ne peut que s’en réjouir. Signe du dynamisme économique de la région, une telle saturation n’en est pas moins préoccupante, tant pour des questions environnementales que pour la qualité de vie des habitants. Nos deux pays sont déjà très liés par un accord de coopération ayant vocation à améliorer la circulation des biens et des personnes entre deux membres historiques de l’Union européenne. Les infrastructures de transport actuelles souffrent d’un trafic toujours plus important. C’est vrai pour l’axe routier, avec les nuisances que cela entraîne pour les habitants, mais également pour l’axe ferroviaire, qui a presque atteint les limites de ses capacités. Bien souvent, mes chers collègues, on peut se rendre compte d’un entretien déficient sur nos lignes SNCF. Nos concitoyens sont par ailleurs de plus en plus nombreux à se rendre au Luxembourg pour travailler tout en vivant en France. Ils pourraient être 135 000 à l’horizon 2030. Avec des flux de marchandises qui croissent d’année en année, la France et le Luxembourg doivent constamment ajuster leurs objectifs. Pour continuer à développer notre économie et nos territoires, il est nécessaire d’investir davantage, afin de créer de nouvelles infrastructures. Investir, signifie créer des emplois et continuer à développer des lignes SNCF entre nos territoires. L’avenant qui nous occupe aujourd’hui concerne l’axe ferroviaire. Le plafond des dépenses précédemment prévues passe de 110 millions d’euros à 220 millions d’euros, et nos deux pays y contribueront chacun pour moitié. membres d’un groupe pro européen, nous ne pouvons que nous réjouir d’une meilleure intégration et d’une meilleure coopération. Cet investissement doit servir à financer un centre de maintenance et l’automatisation de lignes. C’est une excellente nouvelle pour nos entreprises, pour ceux qui empruntent cet axe et pour les habitants de la région.

Il participe en effet à mieux maîtriser le dérèglement climatique. En 2020, le transport routier représentait près de 95 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports dans notre pays. Par ces investissements, nous contribuons à réduire l’empreinte carbone de nos deux pays et à concrétiser nos transitions. Choisir le ferroviaire, c’est participer à préserver l’environnement, mais aussi la santé des habitants de ce couloir. Avec davantage de circulation et un meilleur entretien des locomotives, nous bâtissons dès aujourd’hui les capacités de développement économique de nos deux pays, ainsi que de l’ensemble de l’Union européenne. Cette union est une chance pour notre pays et nos concitoyens. Dans la gestion de ces projets d’infrastructures, il faut nous assurer qu’elle le reste et qu’elle soit créatrice d’emplois. La coopération est fondamentale. Nous devons veiller à la faire prévaloir à toutes les étapes du développement de ces projets. Aucune partie ne doit pouvoir imposer sa volonté à l’autre. Nous ne doutons pas que le Gouvernement y est également attentif. Le groupe Les Indépendants soutiendra donc l’adoption de ce projet de loi de ratification.

il se confronte aussi au défi de la prise en compte de l’impact environnemental du transport, essentiellement routier, pourvoyeur de gaz à effet de serre, de particules fines et d’oxyde d’azote. Dans un tel contexte, il est clair que la mission du protocole de 2018 n’est pas encore accomplie et qu’il faut renforcer la coopération franco luxembourgeoise sur ces enjeux, pour que le report vers le train soit massif, pour que les cars express et le covoiturage trouvent la fluidité nécessaire à leur développement. Ainsi, si l’autoroute A31 nécessite des aménagements dans sa partie sud et centre,

nord de Thionville. À l’instar du Léman Express, il s’agit ici de mettre en place ce qui est, somme toute, un service express euro régional métropolitain.

Les travaux qui sont déjà terminés sont ceux qui étaient les moins coûteux. Le renforcement de l’alimentation électrique subit du retard. Le déploiement progressif des investissements projetés est donc très lent, sans doute pas à la hauteur. Nous avons pris du retard sur nos voisins, notamment en termes de modernisation

d’alerter sur la situation des territoires lorrains transfrontaliers. Près de 117 000 de nos compatriotes qui vivent dans ces territoires travaillent au Luxembourg, et l’on estime

où, par exemple, 30 000 voitures par jour franchissent la frontière à Mont Saint Martin. Il est injuste également dans le financement. En effet, alors que notre pays et ses collectivités formé ces travailleurs et que nous continuons de leur garantir leurs droits au chômage, à l’autonomie, au logement ou encore l’accès aux services publics, les territoires où vivent ces hommes et ces femmes salariés au Luxembourg supportent des coûts sans retirer d’avantages financiers. Malgré ce déséquilibre dans la relation financière franco luxembourgeoise, nous nous obstinons dans le modèle de cofinancement à 50 50. L’avenant, dont il est question aujourd’hui, suit la même logique.

La convention de 2018 devrait être révisée au profit d’un mécanisme de rétrocession fiscale. Un tel dispositif permettrait de respecter de manière effective la libre administration des communes et de mettre fin à leur dépendance au bon vouloir du Luxembourg pour financer ou non tel ou tel projet. La complaisance du Gouvernement avec le Grand Duché me La contribution des frontaliers aux finances publiques du Luxembourg s’élève à plus de 2 milliards d’euros. Ce manque à gagner fiscal pèse particulièrement lourd pour les communes du Nord lorrain. Enfin, j’aimerais également vous exprimer, madame la secrétaire d’État, mon incompréhension face à la décision de ne faciliter le logement des fonctionnaires que dans les 133 communes proches de Genève, avec une indemnité de résidence annuelle de 640 euros. Pourquoi exclure les agents publics des territoires frontaliers du Luxembourg ? Le prix du mètre carré en zone frontalière avoisine aujourd’hui les prix parisiens, cela crée des difficultés pour loger les fonctionnaires locaux. Nos collectivités sont également obligées d’offrir des traitements attractifs pour

à l’instar de nombreux autres élus locaux de bords différents, qu’il est fondamentalement injuste que le Luxembourg ne paie que la moitié de ce projet et qu’aucune négociation diplomatique pour obtenir une compensation fiscale ne soit lancée. Aussi, nous nous abstiendrons sur ce texte.

en 2018, 90 000 Français se rendaient chaque jour au Luxembourg pour y travailler. Cinq ans plus tard, ils sont plus de 120 000 frontaliers à emprunter les routes et le train à destination du Luxembourg, et leur nombre pourrait doubler d’ici à 2050.

La congestion des trafics routier et ferroviaire est une source de difficultés croissantes, quotidiennes, pour les Lorrains qui la subissent : allongement de la durée des trajets, problèmes environnementaux, Cet état de saturation justifie l’augmentation de l’enveloppe prévue par cet avenant. Elle porte à 440 millions d’euros l’investissement de la France et du Luxembourg sur l’axe ferroviaire Nancy Metz Thionville Luxembourg. Nous souscrivons évidemment totalement à ce projet, qui permettra d’augmenter progressivement la fréquence des trains et leur capacité d’accueil, pour atteindre 24 000 places en heures de pointe en 2030.

Ces frontaliers, de plus en plus nombreux, font le trajet quotidiennement entre l’Hexagone et le Grand Duché, ce qui pose d’inévitables problèmes de transport. L’autoroute A31 est régulièrement congestionnée aux heures de pointe, et l’axe ferroviaire Metz Thionville Luxembourg est fréquemment confronté à des incidents, ainsi qu’à des irrégularités de service liées à la saturation de la ligne. Pour répondre à ces difficultés, le Parlement a autorisé, voilà quatre ans, l’approbation du protocole d’accord entre la France et le Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers. Ce texte visait à mettre en œuvre, aux horizons 2024 et 2030, une politique de transports multimodale et concertée entre les deux parties, s’inscrivant dans une perspective de développement durable. Cette politique tendait à répondre aux besoins de mobilité préalablement identifiés, à travers des projets ferroviaires et routiers. Dans le domaine ferroviaire, une série d’aménagements visaient à tripler le nombre de voyageurs quotidiens et pallier ainsi la saturation de l’axe attendue pour cette année. Il s’agissait d’anticiper les besoins de capacité à l’horizon de 2030. Dans le domaine routier, l’objectif était de développer des lignes de cars transfrontaliers, ainsi que le covoiturage, grâce à la création de voies dédiées, de parkings de regroupement et de gares routières. Les infrastructures routières existantes devaient être adaptées en conséquence. Côté français, l’autoroute A31 devait être élargie à trois voies entre le nord de Thionville et la frontière franco luxembourgeoise, et un contournement de Thionville par l’ouest devait être créé. Côté luxembourgeois, le projet prévoyait une troisième voie de circulation sur l’autoroute A3 et l’aménagement de sa bande d’arrêt d’urgence en voie réservée pour la circulation de cars. La solution retenue est donc multimodale, puisqu’elle s’appuie sur les transports collectifs et qu’elle est complétée, sur le territoire luxembourgeois, par le développement de moyens de transport plus propres, comme le vélo électrique. Le coût total de ces travaux était estimé à 220 millions d’euros pour le volet ferroviaire et à près de 20 millions d’euros pour le volet routier, financés à parité par la France et le Luxembourg. Quatre ans après l’adoption de ce premier accord, quel bilan peut on dresser ? Les aménagements ferroviaires prévus pour 2024 ont été réalisés pour une partie d’entre eux, ou sont en voie de l’être pour les autres, avec un léger retard. S’agissant du volet routier, aucune avancée ne s’est concrétisée pour le moment. Une séquence de concertation s’est tenue voilà un an sur le secteur nord du projet A31 , afin d’éclairer l’État dans le choix du tracé pour le contournement de Thionville. Il faudra donc concentrer toute notre énergie dans ce domaine. L’avenant au protocole soumis à notre examen vise à prolonger les objectifs du protocole de 2008, c’est à dire accompagner l’augmentation des trafics entre la France et le Luxembourg en renforçant les mobilités durables. Le Premier ministre luxembourgeois a annoncé en juin 2021 une nouvelle contribution financière de 110 millions d’euros pour les infrastructures ferroviaires d’intérêt commun à la France et au Grand Duché. Cette participation supplémentaire, qui s’accompagne d’une contribution française identique, permettra de compléter le programme d’investissements de l’accord initial par le financement de besoins identifiés à la suite des études de faisabilité pour l’horizon 2028 2030. Deux projets sont envisagés à ce stade : premièrement, la construction d’un centre de maintenance à Montigny lès Metz ; deuxièmement, la conduite d’études sur l’automatisation ou la semi automatisation de la conduite des trains, dont la réalisation sera décidée en fonction des résultats. J’ai pu observer en commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées que certains de mes collègues s’interrogeaient sur la place décisionnelle qu’occupe la France dans cet accord. Je souhaiterais les rassurer en réaffirmant que la France défend ses intérêts dans cette coopération franco luxembourgeoise. Je voudrais rappeler que ce texte est essentiel pour poursuivre l’amélioration de la liaison ferroviaire franco luxembourgeoise et répondre aux difficultés de mobilité quotidiennes rencontrées par nos concitoyens à l’approche de la frontière. En conséquence, je préconise, au nom du groupe RDPI, l’adoption de ce projet de loi, déjà voté par l’Assemblée nationale le 29 juin 2023.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur il y aurait beaucoup à dire sur ces conventions et, plus largement, sur nos relations avec le Luxembourg, tout particulièrement sur le volet mobilité, si important pour la vie de dizaines de milliers de travailleurs frontaliers et de centaines de communes et collectivités. Alors que nous sommes appelés à nous prononcer sur une augmentation des efforts budgétaires pour l’investissement dans les infrastructures de transports qui permettent, comme l’a justement dit et écrit le rapporteur, à plus de 120 000 Français de se rendre au Luxembourg quotidiennement, je suis au regret de vous annoncer que, pour les Lorrains, 100 millions plus 110 millions font moins que 210 millions, comme si deux plus deux aboutissait à trois. Autrement dit, j’estime que notre voisin et ami luxembourgeois ne met pas assez d’argent sur la table. En effet, comment se satisfaire aujourd’hui d’un engagement de 210 millions

Pour nos bonnes relations interétatiques, je comprends que cela ne soit pas indiqué dans l’étude d’impact, mais la vérité est que le Luxembourg fait son marché dans les projets qu’il consent à soutenir. Il refuse d’investir dans le routier et privilégie le ferroviaire au nom, dit il, du développement durable. C’est un argument qui peut s’entendre. Mais comment accepter, par exemple, que ce pays continue de refuser de cofinancer l’achat de nouvelles rames, comme c’est le cas depuis la convention de 2018 ? Je regrette, monsieur le rapporteur, que vous n’ayez pas suffisamment pointé ce problème dans votre rapport, tout comme je m’étonne du manque de données chiffrées. À peine 10 000 des 120 000 travailleurs frontaliers, soit 8 %, se rendent au Luxembourg par voie ferrée. L’objectif est de passer à 15 avec 22 000 passagers en 2030, ce qui nécessite 600 millions d’euros. Pourquoi est ce que cela devrait être essentiellement financé par les collectivités françaises ?

d’augmenter les cadences ferroviaires pour s’approcher du débit d’un véritable RER. Cela nécessite l’éventuelle réalisation de tout ou partie d’une troisième voie. Pourquoi cette option n’est elle pas envisagée, comme pour le Léman Express ?

est facile de calculer que nous en avons plus de 100 000 par la route. Il faut donc s’attaquer d’urgence aux bouchons quotidiens de l’A31, que nous ne connaissons que trop bien avec mes collègues parlementaires lorrains.

Cette mise à contribution des poids lourds pénalisera principalement les flux étrangers, majoritaires sur cet axe, garantira des recettes stables et substantielles pour la région qui lui permettront d’aller sur les marchés obligataires emprunter à long terme dans d’excellentes conditions, et financer ainsi rapidement la réalisation et la modernisation de l’A31, avec, entre autres aménagements, la création de lignes de bus et de covoiturage express. Pour en revenir au texte, comment peut on accepter que le pays qui détient le record du monde du PIB par habitant contribue aussi peu, peu, d’autant plus que cette maigre contribution de 210 millions d’euros sur six ans est à comparer à tout ce que l’afflux de travailleurs frontaliers rapporte à notre voisin ? Prenez ne serait ce que les 800 millions d’euros par an d’impôts prélevés à la source sur les revenus des 123 000

L’effort contributif du Luxembourg, même faible, ne permet donc pas de multiplier les projets, mais devient un simple transfert budgétaire. Il en est de même pour l’État, qui ne flèche pas les recettes vers ce territoire. Tant mieux pour les autres, mais dommage pour le Nord lorrain ! Mes chers collègues, j’espère avoir clairement démontré l’insuffisance de cette convention de partenariat avec le Luxembourg. Il faut intensifier les efforts de l’État et de la région pour

c’est toujours une grande fierté pour une Mosellane de pouvoir s’exprimer devant ses pairs de la Haute Assemblée sur un sujet qui concerne son département. Le débat du jour porte sur de multiples sujets – européen, économique et environnemental –, avec un impact direct sur le quotidien de mes concitoyens, qui manquent d’une solution adaptée à leurs besoins de mobilité. Plus de 120 000 Français travaillent aujourd’hui au Luxembourg, et leur nombre ne cesse de croître d’année en année. Les déplacements ont très rapidement commencé à poser problème sur nos axes transfrontaliers. Aujourd’hui, l’A31, en particulier, cristallise plus que jamais les tensions. Face à une autoroute congestionnée et des lignes ferroviaires saturées, une solution devait être dégagée de manière bilatérale, à la fois pour endiguer ce phénomène et préparer l’avenir de nos échanges avec le Luxembourg. Pour répondre à ces difficultés, le Parlement a autorisé, voilà quatre ans déjà, l’approbation du protocole d’accord entre la France et le Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers. Aux horizons 2024 et 2030, ce texte devait permettre la mise en œuvre d’une politique de transports multimodale et concertée entre les deux parties, à travers des projets ferroviaires et routiers. Avant toute chose, il faut le reconnaître, ce protocole d’accord et l’ensemble de la démarche étaient nécessaires, tant cette question est devenue épineuse. Malheureusement, il faut également admettre que ces efforts sont encore insuffisants face à l’ampleur du problème et aux enjeux. Ainsi, l’avenant au protocole soumis à notre examen vise à prolonger les objectifs de 2018, c’est à dire à accompagner l’augmentation des flux entre la France et le Luxembourg en renforçant les mobilités durables. Dans cette optique, le Premier ministre luxembourgeois a annoncé en juin 2021 une nouvelle contribution financière de 110 millions d’euros pour les infrastructures ferroviaires d’intérêt commun à la France et au Grand Duché. Cette contribution est complétée d’une somme identique par l’État français, mais cet avenant se concentre, malheureusement, essentiellement sur le ferroviaire. Les aménagements ferroviaires prévus pour 2024 sont en pleine réalisation. Je pense notamment à l’allongement des quais, ou à l’aménagement des parkings relais, comme en gare de Thionville. Deux nouveaux projets sont envisagés. Tout d’abord, la construction d’un centre de maintenance à Montigny lès Metz qui permettra d’assurer la desserte de l’axe avec une plus grande fréquence. Ensuite, l’automatisation ou la semi automatisation de la conduite des trains, dont la réalisation sera décidée en fonction des résultats d’études préalables concernant à la fois l’opportunité et l’intérêt d’une telle opération. Ces deux aménagements supplémentaires devraient réduire les nuisances liées aux mobilités ferroviaires des Mosellans vers le Luxembourg. Si le volet ferroviaire commence à produire ses effets, rien ne garantit qu’il soit suffisant pour endiguer les problèmes massifs liés au domaine routier. En effet, comment pourrions nous imaginer un instant que le développement des lignes de cars transfrontaliers et du covoiturage serait suffisant pour décongestionner un trafic de plus de 105 000 véhicules par jour En ce qui concerne l’A31 , serpent de mer des projets de mobilité du Nord mosellan depuis des décennies, sa concrétisation, annoncée par Clément Beaune devant le conseil régional du Grand Est ce vendredi 15 décembre, se fera à travers un plan État région de 1.4 milliard d’euros. Ce sera une véritable avancée. L’option choisie du tunnel profond est sans conteste celle qui produira le plus d’effets bénéfiques. Elle limitera l’impact environnemental le long des vallées de la Fensch et de l’Orne, et évitera de scinder la ville de Florange Pour conclure, malgré ses lacunes évidentes, la signature de cet avenant est une étape indispensable, afin de faciliter la mobilité de nos travailleurs transfrontaliers. Deux points suscitent néanmoins des interrogations fortes l’ambition des actions mises en œuvre et l’investissement du Grand Duché pour les infrastructures routières. En effet, on ne peut que regretter de voir nos partenaires luxembourgeois s’investir si peu dans des infrastructures routières, dont ils sont pourtant les premiers bénéficiaires.

En effet, madame la secrétaire d’État, les efforts de la France pour favoriser le ferroviaire et les alternatives à la voiture en général se heurtent malheureusement encore régulièrement à la réalité de nos territoires. Le ferroviaire ne saurait à lui seul empêcher l’aggravation de la situation routière. Les Mosellans attendent encore du Gouvernement des efforts supplémentaires, et je pense que celui ci l’a bien compris : la signature du plan État région mentionné précédemment et la mise en chantier de l’A31 Dans l’attente des prochaines étapes de ce projet historique, le groupe Les Républicains du Sénat soutiendra cet avenant, qui, à défaut de résoudre à lui seul tous les problèmes de congestion de nos réseaux de transports transfrontaliers, devrait permettre d’amoindrir les effets néfastes de ceux ci dans les prochaines années. La parole

pour soutenir les infrastructures et les services transfrontaliers. La question de la fiscalité ne peut pas être absente du débat. C’est pourquoi nous défendrons un projet de compensation fiscale au profit des territoires.

Un système de compensation aux frontières existe déjà avec Genève, qui reverse directement aux collectivités une partie de l’impôt sur le revenu des travailleurs ; d’autres pays le font également. En cinq ans, le Luxembourg n’a engagé que 25 millions d’euros de dépenses sur des projets de codéveloppement choisis par lui. Cela représente un investissement du Luxembourg sur le territoire français de quelque 35 euros seulement par an et par frontalier. Rappelons que l’inaction a un coût et que ce coût se révélera plus important pour le Luxembourg s’il ne fait rien ou trop peu. Il doit prendre à sa charge une partie du service transfrontalier et faire un effort en matière de fiscalité. Tout en votant le texte, nous continuerons, avec Olivier Jacquin et quelques autres parlementaires concernés par le territoire et la problématique, à nous battre pour aller plus loin et obtenir des mécanismes de reversement local et de compensation. Très

pour. Acte vous est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

pour examiner le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) en matière d’économie, de finance, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dans le texte issu de vos travaux en commission. Le droit français s’enrichit régulièrement de dispositions décidées conjointement avec les États membres. À quelques mois des élections européennes, je suis convaincu que l’Europe apporte du bien à la France et que la France en apporte au moins autant à l’Europe, à condition naturellement que la France joue pleinement son rôle dans la construction européenne. J’estime qu’elle l’a très bien fait ces dernières années, et j’espère qu’elle continuera à le faire. Ce texte doit permettre à la France de disposer d’un droit national conforme aux évolutions législatives européennes récentes. Il aborde un nombre très varié de sujets sur lesquels je ne me prononcerai pas de manière exhaustive à cette tribune ; nous y passerions la nuit ! Je laisserai le débat dans l’hémicycle nourrir les échanges sur la plupart des points qui ont suscité votre mobilisation par voie d’amendement. Je veux néanmoins évoquer dès la discussion générale plusieurs points qui nous semblent revêtir une importance particulière. Sur les plans économiques et financiers d’abord, les dispositions de mise en conformité visent notamment donner leur plein effet à des dispositifs en faveur de la protection des consommateurs, ainsi qu’à préciser les règles applicables aux sociétés, ainsi que différents textes de droit national dans les domaines du droit bancaire, monétaire et financier. Le projet de loi permettra, par exemple, aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de contrôler les obligations prévues par le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs en matière d’information du consommateur et d’accès aux moyens de paiement. Il permet de prêter assistance à la Commission européenne dans le cadre des enquêtes réalisées pour mettre en œuvre le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. En tant que ministre chargé de l’industrie, c’est un point qui me tient particulièrement à cœur : nous ne pouvons pas accepter que des subventions indûment versées dans des États tiers mettent en difficulté nos entreprises nationales. nationales. Le texte adapte ensuite le droit national au nouveau cadre établi par le règlement relatif à la sécurité générale des produits, afin de tenir compte des dispositions du droit de l’Union européenne relatives aux services numériques et aux marchés de cryptoactifs. Il prévoit la ratification de l’ordonnance du 24 mai dernier portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales et procède à des clarifications bienvenues. par ailleurs d’harmoniser les différents dispositifs nationaux en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales avec ceux prévus par le droit de l’Union européenne. Ce texte introduit enfin des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment en droit interne et désigne explicitement l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en tant qu’autorité nationale compétente sur le contrôle des paiements transfrontaliers. Dans le cadre de l’assistance internationale au recouvrement, il offre une extension de la possibilité d’échange d’informations entre les administrations. En matière de transition écologique, ce projet de loi assure l’effectivité du devoir de diligence de certains opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou en service des batteries par la mise en place de contrôles. Il prévoit l’obligation de reprise des déchets de batteries par les distributeurs – ce point est très important – à titre gratuit et sans obligation d’achat de nouvelles batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine. également des dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, notamment la création d’une nouvelle sanction applicable aux importateurs pendant la phase de transition jusqu’au 31 décembre 2025. 2025. Il transpose enfin en droit français la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone, le nucléaire y étant explicitement mentionné.

un point de contact unique est créé en France, le rôle d’Europol est consolidé, les délais de réponse sont raccourcis et les motifs de refus de transmission des informations sont mieux encadrés. Le projet de loi procède à la mise en conformité du code de procédure pénale avec les dispositions européennes relatives au droit d’accès à un avocat et au mandat d’arrêt européen.

En matière sanitaire et sociale, le projet de loi met en conformité le droit national sur les substances à l’état de microplastiques dans les dispositifs médicaux de diagnostic, et il prévoit des dispositions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants.

et de sécuriser l’exercice, par les établissements de l’élevage, des missions qui leur sont confiées en matière de traçabilité des animaux ; cela a fait l’objet d’un débat intéressant en commission. Ces évolutions sont toutes nécessaires dans les différents champs de la vie économique et sociale de la Nation

Cela a permis à la commission spéciale de ne pas légiférer à l’aveugle et de proposer de modifier substantiellement ce texte par l’adoption d’une trentaine d’amendements. J’ai fait adopter

en matière de droit des sociétés à l’article 4 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs ou en matière de droit de la consommation, à l’article 1, qui adapte le code de la consommation au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et à l’article 2, qui adapte ce même code au règlement sur

sur le bloc d’article 21 à 26 ont permis de résoudre des imperfections de rédaction et des lacunes dans la transposition. À l’article 27, relatif aux échanges d’informations en matière de terrorisme, j’ai souhaité sécuriser le rôle du parquet national antiterroriste en tant qu’autorité compétente.

Nous examinerons également deux articles portant sur le droit de l’environnement et le droit social. Le premier, l’article 31, met en conformité le calendrier national d’interdiction des microplastiques avec le calendrier européen, amélioré grâce de précision juridique. Le second, l’article 32, permet aux fonctionnaires de bénéficier du report des congés non pris pour cause de congé familial ; nous étendons ce principe à l’ensemble des congés familiaux, quatre types de congés ayant précédemment

directive. Le Gouvernement aurait pu agir et préparer une réforme structurelle dès 2021, mais il a attendu le dernier moment, c’est à dire l’envoi d’un avis motivé, en septembre dernier, par la Commission. Le Gouvernement a encore attendu la dernière étape avant l’engagement d’un recours en manquement pour soumettre un texte en urgence aux assemblées.

La réforme pose de lourds problèmes de fond et suscite une profonde incompréhension parmi les OPJ et les magistrats du parquet. Et pour cause ! Le Gouvernement propose de supprimer toute possibilité d’audition immédiate des gardés à vue. Si la directive C encadre cette possibilité de comparution immédiate, elle ne l’interdit pas. La commission spéciale a pris ses responsabilités. Elle a remanié l’article 28, afin d’établir une possibilité d’audition immédiate dans les strictes conditions posées par la directive de 2013. Les amendements adoptés sont donc le reflet de notre volonté de concilier, d’une part, le plein respect du droit européen et des droits de la défense et, d’autre part, la préservation de la sécurité publique, qui elle même suppose que nos policiers et nos gendarmes aient les moyens de conduire efficacement des enquêtes pénales.

Seul un des articles du texte initial a été examiné en procédure normale. À l’article 6, nous avons adopté un amendement visant à réduire de neuf mois à six mois le délai d’habilitation demandé pour la transposition du règlement (TFR), qui porte sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs. L’ordonnance concernant le règlement (MiCA) sur les cryptoactifs devant être prise avant le 9 mars 2024, la commission spéciale a estimé qu’un délai de coordination de six mois était suffisant. Nous avons également adopté un article 7 , sur l’initiative du Gouvernement,

au titre II du projet de loi, qui rassemble des dispositions en matière de transition écologique. Le texte opère la transposition de deux axes essentiels du paquet climat européen Ajustement à l’objectif 55 la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), encouragée par la France depuis de nombreuses années, et la refonte du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Seqe UE). Les évolutions apportées par le Parlement européen et par le Conseil sont venues répondre partiellement aux observations formulées par le Sénat, dans un rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que dans une résolution sénatoriale, afin de renforcer l’ambition environnementale de ces réformes. Notre commission spéciale a donc accueilli favorablement la transposition proposée par le Gouvernement ce projet de loi. Nous avons toutefois pointé le caractère incomplet de la transposition proposée. En effet, les dispositions du texte relatives au MACF ne portent que sur la période transitoire de 2024 à 2025, pendant laquelle les importateurs ne seront soumis qu’à une obligation de déclaration de l’empreinte carbone des produits. Par ailleurs, le Gouvernement renvoie à un prochain véhicule législatif la transposition du second marché carbone (Seqe 2), qui concernera le chauffage des bâtiments et le transport routier, ainsi que les émissions des installations énergétiques et de l’industrie diffuse non couverte par le Seqe UE, à partir de 2027. Néanmoins, nous avons adopté sur ces articles de nombreux ajustements juridiques et rédactionnels, afin d’améliorer la qualité du projet de loi. J’en viens à l’article 19, qui prévoit de faire évoluer les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, en application d’un règlement délégué du 10 février 2023. Cet article nous a semblé peu ambitieux au regard de l’exigence de décarbonation de l’économie. En effet, les modalités de calcul envisagées ne reprenaient pas l’ensemble du cadre européen prévu pour l’hydrogène. Or toutes les étapes liées à sa production et à son utilisation doivent être prises en compte. De plus, ses dérivés ne doivent pas être omis. C’est pourquoi nous avons adopté un amendement complétant l’article 19 en ce sens. En l’occurrence, il s’agissait d’appliquer les recommandations proposées par le Sénat, dans le rapport d’information de la commission des affaires économiques sur le volet énergie du paquet Ajustement à l’objectif 55, ainsi que dans la résolution sénatoriale précitée. Enfin, j’en viens à l’article 20, qui modifie les règles d’homologation des tarifs de redevance des concessions aéroportuaires. Notre commission a déploré la méthode employée par le Gouvernement. En effet, le lien entre cet article et l’objet général du texte est ténu, car il n’applique pas réellement le droit de l’Union européenne. La commission souscrit toutefois sur le fond à l’objectif du Gouvernement d’une tarification mieux adaptée à la réalité économique. Elle a donc étendu la suppression du principe de modération tarifaire à l’ensemble des aéroports entrant dans le champ de l’homologation tarifaire par l’Autorité de régulation des transports, dans le cas où l’équilibre économique de l’exploitation est substantiellement modifié. En définitive, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les articles du projet de loi que j’ai évoqués. La parole

Nous avons généralement peu de temps pour l’étudier. Cette année ne fait pas exception. Je tiens à saluer le travail de qualité qui a été fourni par la commission spéciale, tout particulièrement par nos deux rapporteurs, Daniel Fargeot et Cyril Pellevat. Un texte qui met en conformité le droit interne avec le droit européen est d’importance pour un pays membre de l’Union européenne. Le projet de loi Ddadue est un texte structurant pour la société française.

pouvons étudier ce texte ce soir, c’est seulement parce que des règlements, des directives et des actes législatifs délégués ont été adoptés à l’échelon européen. La Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen sont le trio qui négocie des pans essentiels de notre droit. européens et anti européens se dessine très clairement dans plusieurs pays d’Europe, dont certains ont déjà cédé aux sirènes des eurosceptiques et autres nationalistes. Même quelques pays fondateurs se sont laissé séduire. Cela doit nous alerter de nouveau. La vague prend de l’ampleur. Nous devons être conscients, mes chers collègues, que ce qui se jouera l’an prochain pourrait orienter dans les années à venir notre propre droit interne.

ou rend la notion floue, elle nous expose à une difficulté d’application, à une mauvaise transposition et à de possibles contentieux, comme vous nous l’aviez signalé, monsieur le ministre. Là encore, le peu de temps que nous avons eu pour l’étude de ce texte est en partie la cause du problème.

En tant que chef d’entreprise, je considère qu’il faut procéder à une juste transposition de la directive relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées. La parité est un élément essentiel. Nous serons attentifs aux ordonnances que prendra le Gouvernement. L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est également primordial. Ainsi, la transposition de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants est une bonne nouvelle. Je salue d’ailleurs les évolutions proposées en commission spéciale afin de compléter la liste des congés couverts. La partie relative à la transition écologique insère dans notre droit plusieurs sujets majeurs. Les textes verts européens participent à la réalisation de nos De nombreux sujets sont traités dans le texte, mais je retiens particulièrement les évolutions du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et les règles durant la période de transition du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Sur ce point, je sais quelle a été la détermination de la France, lors de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, pour que ce mécanisme soit une réalité. C’est un instrument essentiel pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu’Européens. Enfin, en ce qui concerne le droit pénal, il sera question du mandat d’arrêt européen, et particulièrement du droit d’accès à un avocat. Nous devons nous accorder sur un texte mesuré et applicable.

un travail particulièrement éclairant sur le vaste champ de ce projet de loi. J’associe bien sûr à ces remerciements le président Allizard, qui a su créer les conditions d’un échange dense et constructif,

Ce texte est éminemment technique, mais il recèle plusieurs sujets qui ont appelé plus particulièrement l’attention. Par le biais des amendements que nous avons adoptés, nous avons veillé à améliorer la rédaction du texte et à en renforcer la sécurité juridique.

dans les conditions où nous l’avons fait, car le sujet est d’importance. En 2021, la Commission européenne a mis la France en demeure de réformer la garde à vue, avant d’adresser un avis motivé, dernière étape avant la mise en place d’un recours en manquement pouvant être assorti de sanctions financières.

pour apporter des clarifications aux conditions dans lesquelles la nouvelle procédure de recours à l’avocat pourra être mise en œuvre. La commission a ainsi supprimé les incertitudes et les risques juridiques que posait la rédaction initiale du projet de loi. Elle a également rétabli la possibilité d’une audition immédiate des gardés à vue dans le respect des strictes conditions prévues par le droit européen. Ce projet de loi Ddadue opère également la transposition du paquet climat européen Ajustement à en prévoyant la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et la refonte du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. d’ailleurs noter une vraie cohérence entre les évolutions apportées par la commission et le travail opéré en amont, au Sénat, par le biais d’une mission d’information. J’en viens à un sujet que je suis plus particulièrement, celui de la modération tarifaire appliquée aux aéroports. le rapporteur Cyril Pellevat l’a rappelé, l’article 20 du projet de loi vient aménager ce principe de modération tarifaire, dans un cas particulier, pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession. La commission spéciale, lors de nos travaux, a indiqué souscrire à l’objectif du Gouvernement d’éviter que l’appel d’offres relatif à un aéroport du Grand Ouest – car

Ce texte apporte aussi de nouvelles protections pour les consommateurs, l’article 2, qui adapte le code de la consommation au règlement relatif à la sécurité générale des produits. Ce dernier entrera en vigueur au mois de décembre 2024. Il vise notamment à améliorer les rappels des produits et à renforcer les obligations d’information et de coopération des places de marché en ligne avec les autorités face à la hausse de la dangerosité de certains produits.

qu’il sera difficile pour l’Union européenne d’atteindre ses objectifs environnementaux d’ici à 2030 et appelle les États membres à appliquer davantage les lois existantes et à intégrer le climat et l’environnement dans d’autres domaines politiques.

féliciter que la directive sur le marché carbone, pierre angulaire du Pacte vert, prévoie l’application du principe de pollueur payeur. Toutefois, reconnaissons que le maintien des quotas gratuits dans certains secteurs jusqu’en 2034 est une aberration climatique et économique, dénoncée jusqu’à la Cour des comptes européenne.

Ainsi, la forme n’est pas éloignée du fond. Les principes démocratiques qui nous sont chers sont malmenés par le Gouvernement, qui attend la dernière minute pour poser la question de la conformité du droit français

À l’inverse, nous n’hésitons pas à tordre les dispositions européennes quand elles cherchent à mieux défendre les libertés individuelles, comme dans le cadre du régime de garde à vue. Ces écarts que vous vous permettez par rapport au texte initial et aux dispositions de l’Union européenne révèlent, au fond, la vision que vous défendez pour la France et, à travers elle, pour l’Europe.

d’adaptation au droit de l’Union européenne. Avant les dindes, les Ddadue ! Au delà de l’apparente complexité et technicité que ces mesures revêtent, ainsi que de la faible marge de manœuvre qui nous est laissée à nous, parlementaires, pour transposer le droit européen, nombre de nombre de ces dispositions auront un impact important sur le quotidien de nos compatriotes. Ainsi, leur apport mériterait d’être davantage souligné.

mettant fin notamment à des dérogations à l’accès à un avocat, qui, je le répète, ont poussé la Commission européenne à mettre en demeure la France en 2021, puis à lui adresser, il y a quelques semaines, un avis motivé, dernière étape avant un recours en manquement potentiellement assorti de sanctions financières.

s’est réjoui tant de la suppression initiale du délai de carence, mentionné à l’alinéa 1 de l’article 63 4 2 du code de procédure pénale, que de la possibilité ouverte au procureur

les travaux de la commission spéciale qui ont permis d’étendre le périmètre de l’article 64 du code de procédure pénale, afin de garantir que la renonciation à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue soit consignée en procédure.

Je pense ici aux dispositions bienvenues de transposition du Pacte vert pour l’Europe, permettant la refonte du système d’échange des quotas d’émission de l’Union européenne et la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Néanmoins, nous ne pouvons nous satisfaire de l’adaptation de notre droit national au règlement du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique – autrement dit, les microplastiques. En vertu de notre calendrier d’interdiction nationale des microplastiques, désormais conforme au calendrier européen récemment adapté, les dispositifs de diagnostic des émissions de microplastiques

De la même manière que pour le glyphosate, si elle ne peut se permettre d’avoir une législation plus dure que ses voisins européens, la France doit s’entendre avec eux sur une trajectoire commune de réduction et d’accompagnement planifiée,

les projets de loi présentés sous l’acronyme générique Ddadue, dont le contenu est généralement très aride, visent à incorporer à notre droit national un ensemble de directives et de règlements européens récemment adoptés. Celui que nous examinons aujourd’hui n’échappe pas à cette règle : il transpose plusieurs directives et met en cohérence le droit national avec un certain nombre de règlements portant sur des thématiques techniques au champ très large, puisqu’elles concernent tout à la fois l’économie, les finances, la transition écologique, la procédure pénale, le droit social et l’agriculture. En engageant la procédure accélérée sur ce texte, le Gouvernement démontre sa volonté de satisfaire à ses obligations européennes, afin que la France ne présente aucun déficit de transposition et dispose d’un droit national conforme aux différentes évolutions législatives européennes récentes. Certaines dispositions du texte anticipent même les modifications en cours d’élaboration à l’échelon européen, c’est dire

articles ont fait l’objet d’une procédure de législation en commission le 13 décembre dernier, au cours de laquelle les rapporteurs Fargeot et Pellevat, dont je souhaite saluer le travail, ont proposé de nombreux amendements de précision et de clarification rédactionnelle, mais aussi de coordination. aussi de coordination. Le présent texte comporte de réelles avancées. Je pense à l’harmonisation des différents dispositifs nationaux en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales avec ceux qui sont prévus par le droit de l’Union européenne. Citons également les dispositions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants, notamment l’inscription dans le code général de la fonction publique (CGFP) du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition durant certains congés familiaux pour les fonctionnaires. En matière de transition écologique, des dispositions visent à responsabiliser les opérateurs économiques mettant sur le marché ou en service des batteries. Voilà qui permettra d’encadrer ce secteur en plein essor. dispositions tendent à sécuriser le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs. Sur le plan répressif, le texte introduit des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment en droit interne et désigne explicitement l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme autorité nationale compétente pour veiller au respect des exigences européennes concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. Il prévoit aussi des dispositions relatives à l’échange d’informations entre les services répressifs des pays de l’Union européenne et visant à garantir un accès équivalent des services répressifs de tout État membre aux informations disponibles dans d’autres États membres.

À l’heure où la menace terroriste pèse sur de nombreux États européens et où des cellules s’y développent, cette mesure renforcera la capacité de prévention et d’action de nos services de sécurité. Le Gouvernement, qui a entendu les inquiétudes des rapporteurs, nous a précisé en commission que le parquet national antiterroriste conservera la maîtrise de la diffusion des informations méritant d’être transmises à Eurojust. Consulté par la Chancellerie, ce dernier ne semble d’ailleurs pas souhaiter endosser les missions supplémentaires d’animation et de coordination dévolues au correspondant national, actuellement assurées par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice. Quant à la réforme de la garde à vue, les rapporteurs ont considéré que, en l’état, elle viendrait sérieusement compliquer l’efficacité de l’action des parquets et des officiers de police judiciaire Il est donc important d’opérer un travail d’équilibre entre préservation des droits des personnes gardées à vue et prérogatives des enquêteurs et des procureurs de la République.

en raison de l’éloignement géographique du lieu où [elle] se déroule ». Dans son avis motivé du 28 septembre dernier, la Commission européenne considère que l’expression

Il me semble que ce texte ne tombe dans aucun de ces écueils. Pour cette raison, et parce qu’il nous oblige à l’échelle européenne, les sénateurs du groupe RDPI apporteront leur entier soutien au présent projet de loi. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en cette rare occasion où notre assemblée examine la transposition des directives européennes dans notre droit national, je souhaite mettre en lumière trois points soulevés par ce projet de loi qui exigent une vigilance accrue de notre part. Tout d’abord, j’appelle votre attention sur la proposition de mise en conformité de l’article 31, suscite des inquiétudes en raison de la divergence de calendriers entre la directive RED III et notre législation nationale. L’interdiction des microplastiques dans les dispositifs médicaux de diagnostic soulève notamment des interrogations

De plus, elle suscite des préoccupations sur les évaluations entre instances nationales et européennes, ainsi que sur d’éventuelles pressions de lobbies. Doit on y voir une amorce de renonciation ? Les bénéfices attendus en termes de santé publique, notamment la réduction de l’incidence des diverses maladies, sont clairement démontrés dans l’étude d’impact de la Commission européenne. Il est crucial de le souligner, les avantages économiques des mesures de retrait pourraient atteindre environ 31 milliards d’euros par an, offrant ainsi certaines marges financières au profit de la prévention des maladies

La version initiale de cet article avait le mérite de renforcer l’intervention de l’avocat au stade de la garde à vue, ce moment clé de la procédure pénale, dont l’encadrement souffre d’un retard historique dans notre pays. Cependant, les modifications apportées au texte par les rapporteurs en commission spéciale sont en opposition directe avec cet esprit de progrès. En effet, la formule qui a été choisie permettrait de déroger systématiquement à la présence de l’avocat. Nous ne pouvons pas nous permettre de légiférer sur des sujets si complexes et sensibles dans de telles conditions, vous en convenez vous mêmes, messieurs les rapporteurs. Pour ces raisons, nous voterons contre tout amendement qui aurait pour objet la réduction des droits de la défense du prévenu en garde à vue, notamment ceux qui relèvent de la présence d’un avocat. Enfin, l’article 5 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances des mesures pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées. Nous encourageons

Deux principes entrent ici en confrontation ; des solutions devront donc être trouvées sur cette question. La transition écologique demeure aussi un enjeu central pour l’avenir de notre société. Mon collègue Michael Weber détaillera

rapporteurs ! Malgré les réserves que nous pourrions émettre sur certaines dispositions, l’expérience nous a appris que, dans de nombreux domaines, la lutte contre la surtransposition était un enjeu capital. capital. À cet effet, la procédure de législation en commission a été utilisée pour dix huit articles de ce projet de loi. Sans revenir sur l’ensemble des points évoqués à l’occasion de nos débats, je souhaite toutefois vous présenter quelques dispositions qui ont particulièrement retenu mon attention.

Cette mesure parachève une évolution entamée depuis 2021, visant à prévenir un contentieux européen. Elle semble satisfaisante pour les acteurs institutionnels et économiques. Enfin, en matière agricole, sur l’initiative du rapporteur, les travaux de la commission spéciale ont permis d’améliorer le dispositif sécurisant juridiquement les missions exercées par les établissements d’élevage. Les quatre amendements adoptés en commission tendent à conforter le rôle stratégique de l’ensemble des acteurs de la traçabilité animale.

le Gouvernement a préféré préparer, pendant deux années, à huis clos et sans informer le Parlement, une réforme qui doit désormais être adoptée dans l’urgence. Dans ce contexte, je me joins aux critiques qui dénoncent les conditions d’examen d’une réforme

discutables. Ensuite, ce texte transpose deux dispositions essentielles du paquet Climat européen, notamment le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce dispositif, largement soutenu par le Sénat,

Voilà un véritable signal positif adressé aux industriels qui produisent en France et dans l’Union. Il montre que notre pays s’engage dans sa transition écologique non pas contre leurs activités, mais en valorisant les efforts réalisés par les bons élèves et en luttant contre le risque de fuites de carbone. carbone. De même, l’article 15 adapte au secteur aérien l’extinction progressive de l’allocation gratuite des quotas carbone historique. Cette dernière s’accompagne de l’allocation de quotas pour encourager l’utilisation de carburants durables.

déchets associés ou encore au devoir de diligence des opérateurs économiques. Ainsi, vous l’aurez compris, mes chers collègues, notre groupe approuve ces dispositions tendant à mettre notre droit en conformité avec le droit de l’Union européenne, telles qu’elles ont

Tout d’abord, dans un contexte de crise climatique, il est vraisemblable que la batterie électrique sera amenée à jouer un rôle majeur dans la transition écologique. Toutefois, le marché des batteries comporte encore des zones d’ombre. Nous connaissons le coût environnemental et humain de l’extraction minière de ses composants, à l’instar du cobalt en République démocratique du Congo. Prévu à l’article 10, le renforcement des moyens de contrôle de l’administration, des obligations et des contraintes pesant sur les professionnels qui mettent sur le marché des batteries est donc bienvenu. Nous proposerons d’aller encore plus loin en ce sens, en renforçant les sanctions pesant sur les entreprises qui ne respecteraient pas leurs devoirs de diligence et de précaution. Ensuite,

sur notre territoire, afin de valoriser et recycler les matières premières. En ce sens, l’instauration d’une taxe carbone aux frontières doit permettre de lutter contre les importations et exportations de produits polluants, tout en réduisant la délocalisation des activités industrielles européennes.

De manière générale, on peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’un tel marché carbone, qui prétend répondre à l’urgence climatique grâce aux vertus d’une régulation par le seul marché.

Sans une réglementation contraignante et sans la fixation d’un corridor de prix assurant une certaine stabilité, le marché carbone restera inefficace pour lutter contre les émissions carbone. Pis, il entraînera des effets d’aubaine pour les industries les plus polluantes. En ce qui concerne l’article 20, nous tenons à réaffirmer que nous sommes favorables au maintien du principe de modération des tarifs de redevance aéroportuaire par

Nous comprenons aussi les inquiétudes de certains à propos de circonstances exceptionnelles – une crise sanitaire semblable à celle de la covid 19, ou encore une inflation très importante –, qui pourraient susciter des difficultés pour les aéroports. Néanmoins, la notion trop floue « d’équilibre économique substantiellement modifié source potentielle de contentieux, nous rend perplexes. Nous voterons donc pour l’amendement du Gouvernement, qui tend à maintenir le principe de modération tarifaire. Nous tenons en effet à rappeler que certains aérodromes bénéficient du système dit de la double caisse,

L’article 5 de la directive qui serait transposée dans notre droit par ordonnance au présent article ne peut être inférieur aux règles en vigueur. C’est une avancée bienvenue à mettre au crédit du rapporteur. Cet article 5 prévoit que, au 30 juin 2026 au plus tard, l’un des deux objectifs suivants doit être atteint : au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs pour les membres du sexe sous représenté ; au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs. Ces dispositions concernent les seules entreprises cotées, alors même que, dans les sociétés non cotées et les PME, respectivement moins de 25 % et moins de 18 % de femmes atteignent ces responsabilités. Ces modifications permettent de souligner

Comment ne pas s’indigner que, dans les entreprises du CAC 40, au 1 janvier 2022, les femmes occupent 3,75 % des 80 postes de président et/ou de directeur général ?

Il prévoit ainsi que tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros et qui effectue une première mise sur le marché est tenu de respecter les obligations qui découlent de

et environnementaux inhérents à la mise sur le marché des batteries demeurent, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée. Par cet amendement, nous souhaitons donc couvrir le champ le plus large possible.

est librement fixé par l’autorité de contrôle compétente. Or, si une certaine souplesse doit, en effet, être laissée à celle ci, il semble nécessaire de prévoir un délai maximum.

Je le rappelle, l’objectif de la directive européenne est de réduire les risques sociaux et environnementaux liés au cobalt, au graphite naturel, au lithium, au nickel et aux composés chimiques nécessaires aux batteries. Le présent amendement vise donc à prévoir une application rapide et efficace de la loi. Quel de la loi. Quel est l’avis de la commission spéciale ? Les obligations associées au devoir de diligence sont complexes et nécessitent un effort organisationnel important de la part des opérateurs assujettis. Il est donc préférable de laisser l’autorité de contrôle fixer le délai pour corriger un défaut de conformité, en faisant preuve de pédagogie et de souplesse,

le rapporteur. Le présent amendement vise à étendre l’obligation de contractualisation avec les éco organismes ou avec les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries, en cohérence avec le dispositif existant dans la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques et prévu à l’article L. 541 10 20 du code de l’environnement.

en supprimant l’allocation de quotas gratuits aux unités de chauffage urbain et aux hôpitaux couverts. L’amendement n° 20,

du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières se traduira par une réduction progressive des quotas de carbone gratuits.

? Je ne suis pas favorable au quintuplement des sanctions administratives en cas de méconnaissance des obligations de compensation au titre du régime Corsia, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous avons choisi de calquer le niveau de sanctions sur celui qui est applicable en cas de méconnaissance des obligations au titre du marché carbone, soit 100 euros par tonne. Ensuite, je le rappelle, le niveau d’amende est fixé par tonne de CO2

Nous avons travaillé avec le Gouvernement et le sénateur Vincent Capo Canellas à une nouvelle rédaction, qui permet d’assouplir le principe de modération tarifaire, tout en protégeant les usagers d’une hausse injustifiée. Je me félicite de cette nouvelle rédaction de compromis. La commission émet donc un avis favorable

sans recevoir de compensation. En effet, le Gouvernement a fait des avances, notamment sur les questions de sûreté, qui ne sont toujours pas converties en subventions, alors que le dispositif était, semble t il, dans les tuyaux.

pour les aérodromes dont le trafic annuel dépasse 5 millions de voyageurs. Si l’Autorité de régulation des transports peut fixer certains principes et règles relatifs à la régulation des aéroports figurant dans son champ de compétence, elle doit aussi pouvoir rendre des avis sur les projets

La mission de rendre des avis sur les textes réglementaires, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, garantit la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions, donc l’effectivité de la régulation.

l’égale des autorités indépendantes économiques, en alignant ses compétences sur celles des autres régulateurs sectoriels. Quel

Par définition, la présence de l’avocat en garde à vue est souhaitable. Elle doit être garantie ; en aucun cas, elle ne peut représenter une menace pour la démocratie. Le code de procédure pénale prévoit déjà le report de la présence de l’avocat pour protéger la vie des tiers ou assurer le bon déroulement des investigations urgentes.

de la mesure,

pourra prendre connaissance des procès verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence. En outre, au II, nous précisons le dispositif adopté par la commission spéciale, s’agissant de l’inscription au procès verbal récapitulatif de l’article 64 du code de procédure pénale de l’éventuelle renonciation du gardé à vue à l’assistance d’un avocat. L’amendement

Pour pallier la suppression du délai de carence, le ministère suggère également un recours accru au report de l’assistance d’un avocat pendant douze à vingt quatre heures. Il s’agit pourtant d’une procédure exceptionnelle, réservée à la criminalité organisée…

par les termes « éloignement géographique », la directive ne vise que les territoires d’outre mer et le terrain des opérations extérieures menées par les forces armées.

lorsque l’avocat choisi ne peut être contacté ; lorsqu’il déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures ; enfin, lorsqu’il ne s’est pas présenté dans le même délai.

laquelle permet de déroger temporairement à l’assistance d’un avocat pour mener des investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation de preuves. Par esprit d’efficacité, par pragmatisme, mais aussi par volonté de garantir la stricte conformité de notre droit

une décision écrite et motivée : il devra justifier que l’audition immédiate est, au vu des circonstances de l’espèce, indispensable compte tenu de la géographie et qu’elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’être assisté par un avocat. Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable

Cette disposition me semble pourtant cohérente avec la possibilité, pour toute personne gardée à vue, d’informer tout tiers de la mesure, quelle que soit sa qualité.

intervient à l’expiration du délai de deux heures si l’avocat ne s’est pas présenté. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit la saisine du bâtonnier au bout de deux heures lorsque l’avocat ne peut être contacté, ou a déclaré ne pas pouvoir se présenter, ou encore ne s’est pas présenté.

L’amendement n° 28 vise à permettre à l’avocat qui se présente, alors qu’une audition ou une confrontation a déjà eu lieu, de consulter les procès verbaux afférents.

à la possibilité de commencer les auditions, même si l’avocat ne s’est pas présenté. Sur le fond, comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, les termes de l’avis motivé rendu par la Commission européenne que notre droit soit modifié pour se conformer aux exigences européennes. Je suis, par voie de conséquence, fermement défavorable à l’amendement n° n° 7 tend à modifier les critères permettant d’ordonner le report de l’assistance de l’avocat ou l’audition immédiate de la personne gardée à vue sans son avocat. Ce report se ferait afin de « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » actuellement prévues par le code de procédure pénale, plutôt que dans celui d’« éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale », qui correspond littéralement à ce que prévoit la directive 2013/48/UE,

Le plus tôt sera donc le mieux ! En réalité, nous sommes déjà en retard. Le même rapport sénatorial indique que, si les micropolluants proviennent de plusieurs sources, ils convergent vers les milieux aquatiques. Nous polluons donc notre eau et les espèces qui l’habitent.

plusieurs fois pour inaction climatique. Une fois n’est pas coutume, prenons le risque d’être condamnés pour proactivité climatique. Cela nous changera ! Quel est l’avis de la commission

Merci